Chers collègues, l'ordre du jour appelle le débat sur les défaillances d'entreprises à la demande de la délégation aux entreprises. La parole est tout d'abord à l'orateur de la délégation aux entreprises qui a demandé ce débat, monsieur Olivier Rietman, pour la délégation aux entreprises pour huit minutes. C'est à vous, chers collègues.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La délégation aux entreprises a souhaité associer l'ensemble des sénatrices et sénateurs au débat qu'elle a initié en début d'année sur les défaillances des entreprises. C'est un sujet essentiel car nous devons être conscients de la situation très délicate de nombreuses entreprises et nous mobiliser pour les accompagner dans une période marquée par la guerre commerciale internationale et les incertitudes en matière de croissance en France. Le sujet des défaillances est en réalité multiforme. Il y a tout d'abord le constat chiffré qui est sans appel. La très forte croissance du nombre de procédures collectives a dépassé le simple rattrapage post-Covid. Le nombre de défaillances sur un an était évalué à près de 66 000 en février par la Banque de France et à 68 000 selon Altares. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de 2015, et dépasse très largement le niveau des défaillances qui ont précédé la période de pandémie puisqu'en 2019, on comptait 51 356 défaillances. Enfin, les derniers chiffres publiés par l'Observatoire du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. montre que le nombre d'entreprises entrées en procédure judiciaire a augmenté de 2,3% au premier trimestre 2025 par rapport à 2024 et de 23,8% par rapport à 2019. Nous sommes donc bien loin de la décrue annoncée. Je ne souhaite pas m'étendre sur le sujet de la détection et le traitement des difficultés des entreprises, autre aspect du sujet qui a été largement détaillé par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2024. Ce dernier soulignait que le parcours usagé des entreprises en difficulté demeurait complexe et manquait de lisibilité sur les rôles des différents acteurs et la multiplicité des guichets. D'ailleurs Madame la Ministre, vous y avez fait référence lors de votre audition par la délégation il y a 15 jours. Le médiateur national du crédit et le médiateur des entreprises vous ont remis un rapport proposant des solutions très pragmatiques pour mieux accompagner les dirigeants des TPE et PME. Je souhaite en revanche revenir sur la leçon que nous devons tirer de l'évolution des défaillances. Ces chiffres doivent en effet nous alerter. Pourquoi ? Premièrement parce que la situation d'instabilité causée par l'administration Trump laisse planer une menace dont les répercussions seront importantes pour nos entreprises. Nous avons d'ailleurs entendu les organisations patronales sur ce sujet aujourd'hui même lors d'une table ronde consacrée aux entreprises françaises dans la guerre commerciale. Deuxièmement, si les TPE de moins de 10 salariés représentent 85% des procédures collectives engagées, correspondant à environ 1500 emplois supprimés par semaine, on observe une part croissante des PME et ETI dans les défaillances. Ainsi, la part des PME et ETI de plus de 100 salariés a augmenté de 28% en un an. et le coprésident du métier a depuis longtemps alerté sur la fragilisation des entreprises de taille intermédiaire qui, pour la première fois, ne sont plus aussi résistantes que lors des crises précédentes. Le nombre d'ETI placés en redressement a doublé dans tous les secteurs, de la vente de détail à la construction, en passant par l'aéronautique et les cosmétiques. Or, les ETI sont précisément notre force de frappe en matière de commerce extérieur. Enfin, l'évolution des défaillances dépendra largement des décisions que nous prendrons pour réduire le déficit de la France. La dette publique culmine désormais à plus de 3 300 milliards d'euros et les charges annuelles d'intérêt à 59 milliards d'euros. Alors, quand allons-nous prendre conscience de la gravité de la situation et adopter les bonnes mesures ? Nous ne pouvons plus naviguer à l'aveugle en misant uniquement sur l'augmentation des recettes fiscales provenant des entreprises. Nous avons la responsabilité de les accompagner afin de garantir la résilience du tissu productif français dans une période d'incertitude économique. Remettons au cœur des objectifs la compétitivité. Allianz Strade vient de publier sa dernière étude sur les défaillances d'entreprises à l'échelle mondiale. et a dévoilé ses prévisions mises à jour pour 2025 et 2026. Le groupe estime qu'elles continueront d'augmenter au cours des deux prochaines années comment penser que la France pourrait être épargnée sans réforme structurelle adéquate. Il serait irresponsable de reconduire voire d'aggraver le poids de la contribution des entreprises en 2026, car, je le répète inlassablement, ce sont les entreprises qui créent la valeur et financent les salaires et les politiques publiques. Madame la Ministre, qui a prononcé ces mots ? et cela risque de conduire à une baisse de la rentabilité des entreprises, il faut l'accepter. Qui a appelé à une telle politique de la décroissance ? Ce n'est pas notre collègue Yannick Jadot. Ce n'est pas non plus la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier. Non. C'est votre ministre de tutelle en charge de l'économie et des finances, Eric Lombard. Ce n'est pas acceptable et j'y vois une menace pour les décisions à venir à l'endroit des entreprises. Ne nous trompons pas d'ennemis comme l'a récemment fait Jacques Attali en fustigeant les entrepreneurs. Nous devons au contraire aborder sans tabou les sujets mis sous le tapis depuis trop longtemps, notamment les surtranspositions françaises et la comparaison avec les normes et charges de nos voisins européens. le temps de travail et son coût, les réformes structurelles pour diminuer la dépense publique. Le Sénat, et en particulier sa délégation aux entreprises, sont prêts à se mobiliser pour que les bonnes décisions soient prises afin de redresser les comptes publics sans créer une récession. Afin que les entreprises françaises aient enfin le sentiment d'être accompagnées et soutenues par les pouvoirs publics. Et quand je dis soutenues, je ne pense pas aux aides. Je pense à la capacité de l'État à laisser les entrepreneurs se consacrer en priorité à la création de valeur. La mobilisation devra se faire avec les représentants des entreprises de toute taille. Nous devrons prendre des décisions courageuses et les prendre rapidement. Le temps de la décision politique doit impérativement s'aligner sur celui de la vie économique. Madame la Ministre, je vous remercie pour le dialogue que j'ai l'honneur d'initier ce soir et que mes collègues vont poursuivre au travers de leurs questions. Je forme le voeu qu'ils se poursuivent au-delà de ce débat et avec l'ensemble des ministères concernés. Je vous remercie.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais très sincèrement remercier la délégation aux entreprises de nous permettre d'avoir ce temps d'échange, ce temps de débat sur un sujet très important. Que sont les défaillances d'entreprises ? Vous le savez, un débat constructif commence forcément par des constats partagés à partir de quelques chiffres qui ont déjà été rappelés, mais je voudrais y revenir. Le premier chiffre, c'est évidemment celui des défaillances. 66 000 en 2024, autrement dit, ce sont 66 000 entreprises qui ont connu un jugement d'ouverture d'une des trois procédures collectives, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Le second chiffre à retenir, c'est que parmi ces 66 000 entreprises en défaillance, 32 000, soit environ 48 % employés au moins un salarié. Ce chiffre est à considérer, par ailleurs, à l'aune du nombre de créations d'entreprises chaque année. Depuis 2021, il y a eu plus de 1 million d'entreprises créées, dont une très forte majorité de micro-entreprises, il faut le souligner. Le troisième chiffre que j'aimerais partager avec vous, est celui du nombre d'emplois qui se cachent derrière ces défaillances. Nous l'estimons aujourd'hui à 234 000 contre 151 000 Si ce chiffre alerte, il faut noter qu'environ 70% des emplois amenacés seraient finalement conservés du fait d'un rétablissement ou d'une reprise. L'état des lieux est clair. Notre pays connaît un niveau de défaillance important qui dépasse les niveaux observés avant la pandémie. Mon rôle devant vous ce soir est triple. Le premier est de vous proposer une lecture et une analyse de ces chiffres. Le deuxième, c'est de rappeler combien la compétitivité des entreprises est essentielle. Et le troisième, c'est de vous présenter des solutions sur lesquelles le gouvernement travaille pour enrayer cette dynamique délétère pour notre économie. La première question est évidemment comment expliquerons-nous ce niveau de défaillance. Ce niveau de défaillance que nous observons aujourd'hui doit être replacé dans le contexte du creux exceptionnel des défaillances lors de la crise de la Covid. Entre 2015 et 2019, le nombre de défaillances observées était proche de 56 000 annuellement. Cette baisse drastique du nombre de défaillances s'explique évidemment par l'action du gouvernement et les mesures d'urgence qui ont été mobilisées comme les PGE, le chômage partiel, les fonds de solidarité, l'exonération ou encore le report de cotisation, et ce qui fait que sur les années 2019 et 2020, cette moyenne est passée à moins de 30 000, soit une soit une baisse de plus de 45 %. L'augmentation des défaillances que nous observons aujourd'hui s'explique donc finalement par un effet de rattrapage. Pour autant, notre économie n'est pas grippée et certaines données, non pas conjoncturelles mais structurelles, cette fois, doivent nous encourager. En effet, nous restons aujourd'hui sur une dynamique de création d'entreprises inédites et la création d'emplois dans le secteur privé se poursuit. L'importance de la compétitivité dans notre économie est cruciale puisque finalement nous avons effectivement l'obligation, le rôle de trouver des solutions pour les entreprises qui sont en difficulté lorsqu'elles arrivent aux difficultés mais nous devons effectivement en amont faire en sorte que nos entreprises soient compétitives parce que c'est la compétitivité de nos entreprises qui est essentielle car c'est cette compétitivité qui permet à nos entreprises d'innover. d'investir, de se développer et d'embaucher et de résister également à des effets de concurrence qui peuvent exister au travers les autres pays. Je peux vous assurer ici que le ministre de l'économie et des finances, Eric Lombard, est engagé sur la défense de la compétitivité des entreprises. Pour autant, nos entreprises sont face à une vive concurrence. Elles doivent performer, elles doivent se transformer, elles doivent engager des transitions technologiques, numériques et environnementales. Le gouvernement est pleinement engagé aux côtés des entrepreneurs, qu'il s'agisse des ETI, des PME, des TPE, des entreprises individuelles et des micro-entreprises. Nous sommes là pour les soutenir, les accompagner dans les différentes phases de leur vie. Je veux ici saluer ces entrepreneurs qui sont les acteurs de l'économie, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'économie sociale, et solidaire ou de l'économie conventionnelle, ces entrepreneurs qui assurent la vitalité des territoires et qui génèrent de l'emploi. Je sais aussi, parce que c'est une demande qui revient régulièrement, que nos entreprises ont besoin de lisibilité, de visibilité et de stabilité. Nous devons également nous engager dans une diminution des dépenses publiques pour poursuivre la diminution des prélèvements obligatoires, car ces prélèvements obligatoires aujourd'hui pèsent sur nos entreprises. il ne faut pas oublier, vous l'avez rappelé Monsieur le Président, le poids des normes qui constituent une perte de temps conséquente pour les entreprises et donc une dépense. Et nous en venons à la question de la simplification. Simplifier notre droit, c'est le purger des éléments qui enrayent notre croissance et notre compétitivité et c'est tout l'enjeu du projet de loi simplification de la vie économique qui a été examiné il y a quasiment un an ici et que je continuerai à défendre ce soir à l'Assemblée nationale. Gérer le stock de normes inutiles est une chose, mais il faut également s'attaquer au flux et c'est tout l'enjeu du test PME que nous souhaitons mettre en place et ce combat je le partage avec le président Olivier Ritman. Et il est essentiel pour éviter que ne soit adopté des normes qui apparaissent illusibles pour nos entreprises et qui ont quelquefois un coût disproportionné, notamment pour les plus petites d'entre elles. Nous devons également soutenir notre savoir-faire. Et je le dis très clairement, je recevrai prochainement un rapport de Yves Gégou, ancien ministre, sur le Mad in France pour soutenir effectivement tout ce qui participe à la vie de notre pays, à la vitalité de nos territoires et à des points qui nous sont particulièrement chers. Pour autant, je vous le disais en préambule, notre rôle est également de proposer des solutions pour limiter au maximum ces défaillances et il nous faut structurer notre action pour accompagner les entreprises qui ont des difficultés. Il nous faut mieux prévenir les défaillances et donc agir davantage avant la cessation des paiements, c'est le premier point. Le second, c'est de simplifier la cartographie des outils publics d'accompagnement et le troisième, c'est de repenser le rebond. Le premier chantier est d'inciter les entrepreneurs à agir en amont des procédures collectives. En effet, si 70% des procédures collectives mènent à une liquidation, à l'inverse, 70% des procédures préventives permettent à l'entreprise de poursuivre son activité. L'enjeu est donc de mieux identifier les entreprises à risque. Il existe un dispositif qui est la start-up d'État, signe aux faibles, qui permet d'avoir un certain nombre d'éléments, qui permet d'encourager vers les procédures amiable que sont notamment le mandat ad hoc et la conciliation. Le second chantier est, en mon sens, de simplifier la cartographie des outils publics d'accompagnement. Il existe de nombreux dispositifs et cela ne permet pas aux entrepreneurs de savoir toujours quel est le dispositif qu'ils doivent retenir lorsqu'ils sont en difficulté. Le troisième chantier est celui du rebond. En effet, l'échec entrepreneurial fait l'objet d'une perception particulièrement négative de la société et des entrepreneurs eux-mêmes. Il véhicule une forme d'incompétence et est la source d'une stigmatisation des entrepreneurs. C'est donc un changement culturel qu'il nous faut opérer. Nous avons eu d'ailleurs des travaux qui ont été conduits sur ce sujet dans le cadre d'un groupe de travail guidé par Hélène Bourboulou. Nous avons de la chance d'avoir un certain nombre de dispositifs qui sont à notre disposition et nous ne devons pas repartir d'une page blanche pour construire. Nous pouvons retravailler ces dispositifs et j'espère qu'ensemble, à travers ce débat, nous pourrons esquisser un plan d'action pour répondre à la situation d'urgence que nous traversons. Ensemble, trouvons les moyens pour prévenir, protéger et rebondir. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de deux minutes maximum, y compris l'éventuelle réplique. Le gouvernement dispose, pour y répondre, d'une durée équivalente. Le gouvernement aura la faculté, si le juge est nécessaire, de répondre à une réplique pendant une minute. L'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute. La parole est à notre collègue Franck Ménonville du groupe Union Centrise pour deux minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors que la situation financière de l'État attire l'attention médiatique, celle des entreprises a elle aussi de quoi nous alerter. En effet, la recrudescence des défaillances d'entreprises qui ont dépassé leur niveau de pré-Covid est de plus en plus préoccupante. À la fin février 2025, on dénombrait donc plus de 66 000 défaillances d'entreprises sur les 12 derniers mois, soit une progression en rythme en rythme annuel de 12,5%. Les entreprises de moins de 10 salariés sont particulièrement touchées. Les PME et ETI ne le sont pas moins non plus. Depuis le début 2024, c'est à minima plus de 3 200 postes qui disparaissent par semaine dont plus de 1 200 dans les entreprises de moins de 10 salariés. Aujourd'hui, les secteurs de l'immobilier, de la construction, du transport, de l'automobile sont particulièrement impactés. Les explications sont multiples. Le mouvement de rattrapage post-Covid avec les remboursements des PGE et leurs difficultés de réaménagement l'augmentation des coûts énergétiques le poids du modèle social sur le coût du travail, la prolifération normative, la multiplication des contraintes administratives. Ces entreprises sont pourtant le cœur battant de notre économie. Elles créent de l'emploi, maillent le territoire, génèrent de la croissance, garantissant les savoir-faire et l'innovation. Madame la Ministre, quelles mesures de soutien comptez-vous mettre en œuvre ? Comment mieux anticiper leur défaillance ? Différentes procédures interviennent en amont, telles que le mandat ad hoc qui permet de garder la confidentialité, et c'est important. Il ne représente aujourd'hui que 13% des procédures. Que comptez-vous faire pour favoriser ce type de procédures ? Et enfin, comptez-vous permettre le réaménagement des PGE hors procédures collectives ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Franck Ménonville. Vous m'interpellez sur un certain nombre de points. Vous avez évoqué beaucoup de sujets qui concernent la compétitivité des entreprises elles-mêmes. Effectivement, il nous faut en premier lieu agir sur la compétitivité et finalement diminuer un certain nombre de charges Vous avez posé deux points pour terminer votre intervention. Le premier est comment prévenir les défaillances et le deuxième est finalement comment favoriser un petit peu plus les procédures amiables dont vous avez souligné l'intérêt. En ce qui concerne la prévention des défaillances, il existe un certain nombre de dispositifs aujourd'hui. Un premier qui est celui qui est le plus connu, qui s'établit au niveau du département, au travers notamment notamment des préfectures, et le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises, le co-défi, qui rassemble un certain nombre d'acteurs sur l'autorité du préfet, qui a pour objectif de dépister les entreprises qui présentent des risques de défaillance. L'ADFIP utilise un produit développé par la start-up d'État Signeaux faibles qui permet de consulter un certain nombre d'informations en matière d'effectifs, de ratios financiers, d'éventuels impayés et qui permet d'accéder chaque trimestre à une liste d'entreprises présentant un risque de défaillance à 18 mois. Le codifié échange ensuite avec un certain nombre Environ 40% des entreprises suivies par les commissaires aux restructurations à la prévention des difficultés des entreprises ont été identifiées grâce à signaux faibles. Je pense qu'effectivement tout ce qui permet d'identifier permet d'anticiper et participe à aider. Comment favoriser les procédures amiables ? Il nous faut donner plus de force effectivement à tout ce qui concerne le mandat ad hoc et la conciliation. Je rappellerai que les procédures préventives permettent d'éviter un basculement en procédures collectives. 70% des procédures préventives permettent permettent de poursuivre l'activité. Effectivement, vous avez raison, il nous faut favoriser ces deux procédures amiables. Merci madame la ministre. La parole est à notre collègue Fabien Gay du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Canachy. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre et chers collègues. Bon, il y a deux façons d'aborder ce débat et je remercie le président de la délégation aux entreprises de l'avoir posé. Il y a des défaillances d'entreprises et c'est réel dû aux questions de marché, à la guerre commerciale, au tarif douanier, au prix de notre énergie. C'est vrai et il nous faut traiter ces questions. Et après, il faut aussi se dire y a des entreprises et un patronat qui organisent eux-mêmes la défaillance de l'outil industriel et la délocalisation – oui, vous ne voulez pas l'entendre – et la délocalisation d'un certain savoir-faire en France. 300 plans de licenciement, 300 000 emplois menacés ou supprimés. Je ne suis pas venu vous parler d'ArcelorMittal, Michelin, Auchan. Certains de mes autres collègues vous en parleront. Moi, j'étais hier dans le gare. J'ai été voir une PME, ça s'appelle la verrie du Languedoc. 164 salariés et 100 sous-traitants. Et c'est un sous-traitant quasi exclusif de l'usine Perrier à côté. Cette entreprise, elle est détenue depuis 2011 par Owel-Illinois. Elle n'a aucun problème financier. Leur bénéfice l'an dernier, c'est encore plus 7% par rapport à l'année d'avant. Mais ils ont décidé une stratégie financière, c'est de supprimer 500 emplois et de fermer notamment cette verrie. Et ça va avoir une conséquence, c'est que Paris ne pourra plus embouteiller, ou en tout cas pas dans un circuit court, et on va perdre un savoir-faire. Voilà le réel aujourd'hui. Et cette même entreprise, elle a touché 15 millions d'argent public en cinq ans. Et le réel, c'est qu'elle ne veut pas investir dans le nouveau four, qu'il va falloir, dans les 18 prochains mois, vers à 60 millions d'investissements. parce qu'on n'a jamais conditionné les aides publiques à la question de l'outil industriel. Donc je pose une question. Est-ce que nous allons continuer et le ce gouvernement à avoir les bras ballants sur cette question de stratégie purement financière qui casse nos savoir-faire et notre industrie en France ? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je voudrais d'abord souligner l'engagement d'un certain nombre d'entreprises pour continuer à innover, investir, se transformer et embaucher. Pour autant, le gouvernement regrette profondément la décision de l'entreprise dont vous avez fait état, l'usine de Verri de Vergès, à proximité de Perrier, qui a décidé effectivement d'organiser un projet de réorganisation s'inscrivant dans un contexte économique et financier difficile lié à une baisse structurelle de la consommation des boissons telles que les eaux minérales, le vin et la et la bière, effectivement. Cette réorganisation est présentée comme indispensable par le groupe ONC Illinois afin de conserver sa très forte implantation en France avec neuf sites à ce jour et 2000 emplois correspondant auxquels il faut ajouter plusieurs centaines d'emplois de sous-traitance. Vous dire également que le gouvernement et les services de l'État sont pleinement engagés pour un, vérifier la qualité du dialogue social avec les organisations syndicales et le respect de la procédure d'information et consultation du comité social et économique, vérifier également la qualité des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi, tenant compte des spécificités de chacun. des sites et de s'assurer de la qualité des résultats des actions menées pour rechercher un repreneur pour la verrie de Vergès dans le cadre de la loi Florence et pour une durée de quatre mois. Vous direz effectivement que pour un certain nombre d'entreprises Des solutions avec des repreneurs existent. Nous en avons la preuve avec la Fonderie de Bretagne pour lesquelles un repreneur a été trouvé il y a quelques jours. C'est derrière plus de 250 emplois. Donc des reprises existent. Il faut effectivement se mobiliser pour trouver au mieux un repreneur pour cette entreprise. En tout cas, le gouvernement est complètement engagé dans ce sens. Merci Madame la Ministre. La parole est au président Guillaume Gontard du groupe Ecologistes Solidarité et Territoires pour deux minutes. Merci Monsieur le Président. Vancorex, ArcelorMittal, Michelin, les Fonderies de Bretagne, General Electric, Photowatt, ça vient d'être rappelé. Dans toute la France, les sites industriels ferment avec leur lot de licenciements, de pertes de savoir-faire et de territoires meurtris. Et pendant que vous parlez de réindustrialisation des activités aussi stratégiques que l'acier, la chimie, les pneus, les éoliennes, les panneaux solaires sont liquidés les unes après les autres, à chaque entreprise qui ferme, c'est toute une filière qui se retrouve en difficulté via des effets dominos. Certes, la compétition asiatique, la guerre commerciale américaine et les prix élevés d'énergie expliquent en partie les difficultés actuelles. Mais la plupart de ces entreprises sont rentables. Rentables et leur choix ont pour seul objectif de rémunérer encore plus ses actionnaires, qu'il s'agisse de M. Mittal, déjà riche de 18 milliards de dollars, ou de fonds d'investissement comme BlackRock, à la manoeuvre chez Michelin et General Electric. Face à cette rapacité qui détruit notre souveraineté industrielle, que fait l'État ? Quand il faut subventionner des nouvelles usines, la recherche ou la décarbonation, il est effectivement au rendez-vous, souvent sans aucun contrôle sur l'usage des aides. En revanche, quand il faut sauver ces entreprises, il devient tout à coup impuissant, comme si les délocalisations et les licenciements étaient des fatalités divines. L'État peut pourtant agir. Par exemple, en nationalisant des activités stratégiques, nous avons su le faire avec succès pour les chantiers de l'Atlantique, les câbles sous-marins d'Alcatel. Pourquoi donc pas pour d'autres ? Lorsque les projets de reprise en coopérative par des salariés qui maîtrisent et aiment leur travail existent, pourquoi ne sont-ils jamais retenus et accompagnés ? Madame la Ministre, vous venez encore de le décrire, la destruction créatrice que vous encouragez détruit toute notre industrie et l'intelligence artificielle ne remplacera jamais les savoir-faire humains perdus au passage. Qu'attendez-vous pour agir ? n'y a pas de fermetures. Pour autant, je voudrais quand même redonner quelques chiffres faisant état de la réindustrialisation. 2024 a marqué une année de continuité dans la réindustrialisation au niveau du pays. La hausse se poursuit et la dynamique qui a été enclenchée en 2022 se confirme tout en prenant en compte des difficultés conjoncturelles. C'est vrai. Avec 89 ouvertures nettes de sites au total en 2024, on comptabilise 450 ouvertures nettes depuis 2022. On reste donc sur un chiffre et c'est à souligner parce qu'il y a quelques mois les prévisions n'étaient pas sur cette ligne dans la bouche de certains commentateurs. Ce solde positif, il faut aussi le mettre en avant parce qu'il nous encourage à tenir bon, à continuer à soutenir les entreprises. à persévérer, accélérer sans nier les difficultés. Il ne s'agit pas de ne pas les voir, mais il ne faut pas non plus céder à la fatalité. Les chiffres nous montrent également une réalité. La situation est très contrastée dans le secteur industriel. Là où les secteurs énergaux intensifs souffrent, les industries vertent également. et l'agroalimentaire font des scores admirables. Les industries vertes, je le redis parce que je ne l'ai pas forcément bien dit, et l'agroalimentaire font de très bons scores. Il n'a cependant échappé à personne que la conjoncture actuelle est difficile mais encore une fois il n'y a pas de fatalité. Il nous faut soutenir nos entreprises, les accompagner, actionner tous les leviers nécessaires pour faire en sorte que nous ayons une reprise de la compétitivité et assurer leur prospérité économique. Il y a le projet de loi simplification qui va apporter un certain nombre de réponses en matière de ZAN, de raccordement, en matière de coûts de l'énergie. Il y a tout ce qui concerne le plan d'urgence au niveau européen et il est important que nous ouvrions également le débat sur le coût du travail et qu'on reprenne dès que possible la réflexion sur la baisse des impôts de production pour soutenir la compétitivité de de nos entreprises. Oui, merci Madame la Ministre. Moi je vous posais une Oui, merci Madame la Ministre. Moi je vous posais une question sur la stratégie justement du gouvernement face à cette désindustrialisation qui est effectivement en marche et surtout de quelle manière vous allez réellement agir puisque tous les outils qui sont à votre disposition vous les refusez à chaque fois que ça soit des associations temporaires, que ça soit des aides à des coopératives, que ça soit de l'accompagnement et surtout du travail avec les collectivités. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Est-ce que vous souhaitez répliquer ? Vous avez une minute. Merci Monsieur le Président. Alors juste vous dire que puisque vous avez évoqué à deux reprises la situation des SCOP. En qualité de ministre de l'économie sociale et solidaire je me suis intéressée à ce sujet. Effectivement nous avons aujourd'hui une difficulté pour que des structures comme les SCOP ou les SIC puissent je dirais disposer d'outils de financement équivalents à ceux qui existent pour l'économie traditionnelle. Je vais vous prendre par exemple l'exemple du prêt transmission que propose BPI France. C'est un prêt transmission qui est adapté et qui nécessite que la structure qui reprenne dispose de trois années d'ancienneté. Donc effectivement une scope ou une cycle qui est constituée pour reprendre une entreprise ne peut pas bénéficier de cette ancienneté. Donc nous travaillons avec BPI France en ce moment pour trouver une solution. Nous avons d'ailleurs, je sors de la conférence des financeurs de l'économie sociale et solidaire où nous cherchons un certain nombre d'outils pour organiser un financement pour ces structures. Merci madame la ministre, merci merci monsieur le Président. Vous avez la possibilité de répondre pendant une minute, non ? Très bien. La parole est à notre collègue Marion Canales du groupe socialiste écologiste et républicain pour deux minutes. C'est à vous cher collègue. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Au champ Valet-Au-Vaut-Corex, il y a bien sûr ces fermetures et plans sociaux catastrophiques des grands noms qui attirent l'attention. Dans le Puy-de-Dôme, mon département comme ailleurs. Mais ces annonces relèvent souvent plus de la décision stratégique, ça a été rappelé par mon collègue Fabien Guay, que de la défaillance à proprement parler. J'en profite néanmoins pour parler de la décision scandaleuse du groupe au champ. de fermer le magasin des quartiers nord de ma ville à Clermont-Ferrand parce que c'est un choix stratégique de la famille Muliaise, propriétaire d'Auchan qui condamne des dizaines de salariés alors que, chacun le sait, 10% des dépenses alimentaires et d'équipements des Français aboutissent dans la famille Muliaise. Ce soir je veux parler parce que c'est le débat qui nous occupe par la délégation des entreprises. Des vraies défaillances et des plus petites entreprises sont celles qui le subissent le plus, le président Reitman l'a rappelé. 31% entre octobre 2023 et 2024 dans le Puy de Dôme et c'est un sujet qui nous tient tous à cœur et qui se déroule souvent plus à bas bruit. La loi a confié au tribunal de commerce un rôle de prévention et un rôle actif dans la détection des difficultés des entreprises le plus en amont possible afin de les aider à les surmonter. Pousser la porte du tribunal de commerce, c'est faire confiance à des femmes et des hommes qui, comme les chefs d'entreprise en difficulté, sont eux aussi issus du monde de l'entreprise. Mais alors que le nombre de salariés dont l'emploi est menacé par une défaillance de l'entreprise a triplé dans mon département, Clairement vers Métropole a par exemple pris la décision de ne pas rester sans rien faire, donc une collectivité, et de venir conforter ce rôle de prévention assumé par le tribunal de commerce en créant un dispositif permettant d'intervenir au stade de la procédure amiable. La métropole a signé une convention, créé un fonds et délivre une subvention à l'association des justes et enceintes. Justes consulaires du Puy-de-Dôme pour les accompagner. Chaque année, c'est plus d'une douzaine d'entreprises qui est accompagnée pour ne pas venir gonfler les chiffres. La région Ile-de-France a initié le chèque prévention. Madame la Ministre, vous nous l'avez dit, il y a des initiatives en matière de prévention mais les chefs d'entreprise ont besoin certes d'être identifiés mais d'être aidés avec de l'argent. Est-ce que l'Etat va se saisir de ce type d'initiative des collectivités locales pour les généraliser et passer de la culture de la défaillance à une culture de prévention et du rebond ? Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice Marion Canales. Vous évoquez finalement un certain nombre de dispositifs qui existent et qui ne donnent pas forcément de lisibilité ou de clarté. pour franchir la porte du tribunal de commerce comme vous l'indiquez. Effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire et je pense qu'il nous faut gagner en lisibilité pour faciliter l'accès des entreprises et pour savoir finalement à quelle à quelle porte elles doivent frapper. J'étais la semaine dernière dans la Loire, j'ai pu échanger avec le préfet, avec les services de la préfecture qui ont organisé un système, un dispositif sur la prévention des difficultés en associant l'ensemble des acteurs, à la fois les acteurs publics publics et également des acteurs privés, sur le modèle du comité qui avait été créé durant la crise de la Covid, la crise sanitaire et la crise économique. Ils ont maintenu un dispositif qu'ils appellent les rencontres économiques où ils participent à avoir une attention particulière sur tout ce qui est défaillance d'entreprises. Nous avons effectivement en France les conseillers départementaux aux entreprises en difficulté, les commissaires à la restructuration et la prévention des risques, le CIRI. Effectivement, ça n'est pas toujours facile pour les entreprises. Je pense qu'il nous faut avoir une porte d'entrée unique et ce sera un moyen pour mieux accompagner les entreprises et pour probablement aussi mieux les engager dans les deux dispositifs de procédures amiable pour préparer. delà de rechercher des dispositions en matière de soutien financier, il faut travailler sur la compétitivité des entreprises en amont pour faire en sorte que nos entreprises sont encore plus compétitives, arriver à diminuer les prélèvements obligatoires, arriver à diminuer également le coût du travail pour que nos entreprises puissent embaucher embaucher plus facilement et être compétitives par rapport notamment en comparaison avec ce qui peut exister dans d'autres pays et je pense que c'est l'élément essentiel. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Jean-Luc Brault du groupe Les Indépendants, République et territoire pour deux minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président Olivier Rettman, mes chers collègues. Habituellement, quand le bâtiment tousse, c'est l'économie toute entière qui s'arrume, aujourd'hui le bâtiment est grippé, complètement grippé, mes chers collègues. Alors, j'ai deux minutes pour vous parler des défaillances d'entreprises, Madame la Ministre. Il me faudrait deux semaines pour en parler mieux. Empilement de normes sur transposition européenne, concurrence des loyales au sein de l'Union, délai et charges administratives où en est la simplification, accès aux crédits bancaires, agissement et temps de réaction des mandataires liquidateurs. Dernier exemple, tendable ce matin dans mon territoire, le Loir-et-Cher, à l'occasion d'un échange avec un équipementier de la SNCF. 600 salariés, 600 salariés, qui me dit Jean-Luc, dans le nord de la France, je ne citerai pas le nom, j'ai mis deux ans et demi pour avoir un permis de construire, deux ans et demi. En Espagne, il y a six mois, j'ai mis cinq mois pour conclure un permis à Barcelone. et pour pouvoir construire cette usine. Il y a encore deux ans dans notre pays, mes chers collègues, c'est si vous ne tombez pas sur un triton doré ou un papillon azuré. Je n'ai rien contre la biodiversité, au contraire, mais vous avez compris l'idée. Bref, Madame la Ministre, à l'heure où on arrête des chantiers sur chantier, dans le centre de la France aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, qui pèse quand même 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chantier dans le centre de la France, 60 millions d'euros, vient d'être arrêté ce matin définitivement. 60 millions d'euros. Donc où l'immobilier peine à redémarrer ? Où le nombre de restaurants déposent le bilan sans compter ? On a même aujourd'hui des boulangeries qui mettent la clé sous la porte. Nous devons nous mobiliser. Nous avons déposé un texte sur la simplification de la vie économique, il y a plusieurs mois, qui a été voté à l'unanimité. et notamment sur les syndics et sur les mandataires liquidateurs qui font beaucoup de mal dans le cadre des dépôts de bilan et qui font traîner les affaires afin de se servir et de liquider la trésorerie de l'entreprise en difficulté. La question autour du 1er mai aujourd'hui n'est pas le sujet de ces débats, mais n'est-il pas révélateur ? Ne faut-il pas enfin acter une révolution culturelle de l'entrepreneuriat, madame la ministre ? Merci, cher collègue. La parole est à madame la ministre pour deux minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Jean-Louis Brault. Effectivement les entreprises du BTP ont été fortement impactées par les différentes crises et notamment récemment dû à un certain nombre de facteurs. Je pense à tout ce qui est augmentation des taux des crédits immobiliers aux conditions d'octroi des crédits par les banques et à la diminution notamment de la construction qui a un impact direct même si Le marché de la construction neuve diminue, même si de l'autre côté, tout ce qui concerne la rénovation énergétique à vocation accroite, il n'en demeure pas moins que cela a un effet. Et nous devons soutenir au mieux, faire en sorte que le logement reparte, que la construction reparte. Je pense que c'est un élément très important. Deuxième point, il nous faut poursuivre toutes les mesures de simplification dont vous avez fait état. la situation du projet de loi simplification de la vie économique que nous examinons actuellement à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de mesures favorables à la simplification de l'accès à la commande publique pour les entreprises en haussant notamment le seuil de 40 000 à 100 000 euros ce qui va faciliter pour notre très petites entreprises et PME, l'accès à la commande publique. Je pense également à d'autres mesures de simplification qui sont à l'étude au travers les groupements momentanés d'entreprises qui sont un dispositif très intéressant pour les entreprises mais dans la mesure où il y avait une situation de responsabilité solidaire et indéfinie des membres de ce groupement, finalement ce dispositif n'était pas retenu. proposition pour supprimer cette responsabilité solidaire d'un groupement d'artisans ou une PME dans le cadre de marchés de moins de 100 000 euros. Il y a la simplification de l'accès au label RGE également qui est porté par le ministère du logement. Juste vous dire que puisque vous évoquez la situation des restaurants, je lance le 13 mai prochain les assises de la restauration et des métiers de bouche pour travailler avec ces acteurs toutes les situations avec des impacts conjoncturels et structurels. Et juste dans la simplification, je dirai tout à l'heure. La parole est à madame Brigitte Hibert du groupe Les Républicains pour deux minutes. Merci Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre et mes chers collègues. Les chiffres et des défaillances au premier trimestre montrent que les pays de la Loire figurent parmi les régions les plus touchées avec une augmentation de 28%, soit 924 procédures supplémentaires. Dans ma région, 28% des salariés travaillent dans une ETI contre 25 au niveau national. Les ETI attendent une réelle simplification de toutes les procédures. Le programme étincelle est donc plutôt bien accueilli par le milieu économique, car il permet de lever certains freins administratifs pour le bon fonctionnement de nos entreprises. Cela va dans le bon sens et tout ce qui contribue à simplifier la vie de nos entreprises, de nos entrepreneurs doit être encouragé. Cependant, certains freins demeurent et notamment dans l'eligibilité à ce programme. Au sens de l'INSEE, une PME française compte entre 10 et 250 salariés, en deçà, c'est une TPE au-dessus, c'est une ETI. Le critère d'éligibilité au programme étincelle, lui, intègre les PME entre 60 et 220 salariés. Ma question est donc simple. Pourquoi imposer un seuil de 60 ? Pourquoi imposer un plafond de 220 salariés ? Et pensez-vous généraliser ce programme qui aujourd'hui ne profite qu'à trop peu d'entreprises. Élargir le champ des bénéficiaires permettrait de lever des freins pour beaucoup plus d'entreprises et de redonner un élan à l'industrialisation de notre pays. Je vous remercie. Merci cher collègue, la parole est à Madame la Ministre la question de la simplification, vous dire ici, et c'était un point que je voulais aborder, que j'ai engagé une simplification à la fois sur l'aspect législatif au travers du projet de loi simplification, mais également à côté sur tous les modes opérationnels, je peux vous annoncer que lundi matin j'ai fait un point et que sur les 1800 SERFAs que nous avons dont 535 sont sur le volet du monde de l'économie, 535 dépendent du ministère de l'économie et des finances, 115 sont supprimés depuis lundi. Voilà, c'est 115 SERFAs en moins et c'est 450 000 téléchargements qui existaient par an pour ces SERFAs que n'auront plus à faire les entreprises. Donc je le dis, c'est un élément qui va dans le bon sens. Vous évoquez le programme Étincel qui a accompagné près de 200 PME depuis son lancement en 2023 un objectif de 500 d'ici 2027. Ce programme propose un accompagnement effectivement individuel sur mesure pour lever un certain nombre de freins et faire grandir les PME en ETI. Véritablement ça s'adresse à cette cible de PME pour les faire évoluer vers les ETI. C'est un dispositif assez souple pour permettre à une grande diversité d'entreprises de candidats et laisser le choix à la DGE de se prononcer à partir d'un panel représentatif. Véritablement, ce programme a été pensé pour valoriser les pépites de nos territoires. Mais encore une fois, je vous le dis, il est souple et il s'adresse véritablement pour faire évoluer nos PME vers des ETI. Vous avez d'ailleurs dans votre département des entreprises qui en ont bénéficié. Je pense au groupe ABCM, Arcade, Cycle, Rimbaud, Clean, CELS. Voilà, c'est important. Les critères de sélection, comme je vous le disais, sont assez souples. Les appels à manifestation d'intérêt de cette année sont terminés depuis le 28 mars 2025. Le lancement de la cinquième promotion se fera donc le 16 mai En tout cas, encore une fois, si vous avez des entreprises qui souhaitent en bénéficier, je vous invite à vous rapprocher de la direction générale des entreprises. Merci Madame la Ministre. vous avez 36 secondes, d'accord. La parole est à notre collègue le président François Batria du groupe rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour deux minutes. Merci monsieur Merci monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. J'imagine que les questions cet après-midi vont être pour la plupart redondantes. Néanmoins, si personne ne nie si les difficultés des entreprises et le nombre de faillites d'entreprises, de dépôts de bilans par ailleurs, personne ne peut nier non plus l'effort qu'ont fait les gouvernements successifs ces dernières années pour faire de la politique de réindustrialisation une véritable priorité qui a porté ses fruits. Alors on peut porter un schéma dramatique qu'on peut dramatiser à l'extrême. La vie des entreprises a toujours été faite d'entreprises qui se créent, qui disparaissent. C'est la vie des entreprises, il y en a toujours eu. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire dans ce pays. Pendant la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place de nombreux dispositifs exceptionnels, tels que les fonds de solidarité, les frais garantis par l'Etat, les exonérations de charges. Personne ne le nie, tout le monde les demandait aujourd'hui. Mais autant d'aide qu'il y a aujourd'hui, qui ont permis de préserver l'activité de centaines de milliers d'entreprises et de sauver notre économie. Ces dispositifs sont plus à l'ordre du jour. Certaines structures déjà fragilisées rencontrent des difficultés de trésorerie, et vous l'avez dit, l'effet de rattrapage intervient aujourd'hui. Ce sont surtout les petites entreprises, celles qui sont les plus exposées au potentiel hausse de droits de douane, qui font face à des pressions considérables aujourd'hui. Je pense en particulier dans mon département, une entreprise de sidérurgie baltique était un fleuron de la métallurgie de fabrication de tubes en acier, en particulier pour centrales nucléaires dont une historique était située à Montbar et qui a été victime d'une liquidation judiciaire ordonnée le 4 février. par le tribunal de commerce de Dijon. C'est 130 personnes qui risquent de se retrouver sans emploi. Et j'ai entendu aujourd'hui que pour trouver un repreneur c'est difficile. Cela marque la fin d'une époque mais toujours est-il que cet exemple s'inscrit malheureusement et vous l'avez dit parmi tant d'autres. Par ailleurs la guerre commerciale hasardeuse importée par l'administration de Donald Trump engendre aujourd'hui beaucoup d'incertitudes pour le tissu d'entrepreneurs français. Or, que ce soit dans le secteur des produits chimiques, des produits cosmétiques, des parfums, de l'aéronautique ou encore le secteur viticole, nous exportons de nombreux produits issus de notre savoir-faire français. Si nous n'agissons pas dans ces secteurs, Nous serons fortement impactés. Demain, ce seront d'autres acteurs qui prendront leur place avec des groupes étrangers massivement subventionnés, parfois moins soucieux de nos standards et surtout environnementaux. Vous avez déjà, Madame la Ministre, évoqué le travail qui est fait, les pistes que vous envisagez et les mesures qui ont été prises qui portent leurs fruits. Il reste que maintenant, peut-être, je vous demanderai quelles sont les mesures encore plus de simplification qui permettent aux entreprises de pouvoir poursuivre leur activité. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président. La parole est à Madame la Ministre pour deux minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur François Patria. Vous avez évoqué à juste ces titres, et j'avais eu l'occasion de le faire aussi, je dirais la réindustrialisation qui a débuté, je rappelle parce que c'est important, Avec 89 ouvertures nettes de sites au total en 2024, c'est depuis 2022 450 ouvertures nettes. Et c'est vrai qu'il nous faut parler effectivement des défaillances d'entreprises parce qu'il y en a, mais il faut également les remettre à côté avec ces ouvertures nettes. Vous évoquiez l'impact des droits de douane, et effectivement, cela aura probablement un impact. Cela crée en tout cas de l'incertitude actuellement parce que même s'il y a eu une suspension qui a été décidée par Donald Trump par rapport à l'augmentation de 20% des droits de douane qui étaient prévus, c'est une mesure d'apaisement mais il en demeure pour moi que ça crée un moment d'incertitude pendant 90 jours et que par ailleurs il y a tout de même des droits de douane qui ont augmenté de 10% sur un grand nombre de produits et même 25% sur tout ce qui est acier, aluminium, automobiles et produits dérivés. il nous faut utiliser ce moment pour établir un rapport de force pour emmener à la discussion et ça de manière collective, de manière unie au niveau européen. En tout cas, je pense que le monde économique s'est très vite réjoui que l'Europe avait parlé d'une voie unie, collective et sans qu'il y ait deux pays qui partent de manière isolée. Vous demandez un certain nombre de mesures de simplification. Nous en avons qui sont engagées au travers le projet de loi simplification de la vie économique, à la fois sur la commande publique, pour faciliter au travers les artisans d'accéder à la commande publique, pour faire en sorte que les startups innovantes également bénéficient de seuils différents. Nous avons des mesures dans le projet de loi simplification de la vie économique à destination des commerçants, notamment en travers tout ce qui concerne les baux, commerciaux pour faire en sorte que 2 milliards d'euros de trésorerie aillent aillent vers les commerçants par la mensualisation du loyer au lieu et place de la trimestrialisation et la limitation du dépôt de garantie à un mois. Il y a également des mesures à destination des TPE dans ce projet de loi simplification de la vie économique également. Merci madame la ministre. La parole est à notre collègue Philippe Grosvalet du groupe du Rassemblement démocrate et social européen. Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, en 2024, 67 830 procédures de défaillance d'entreprises ont été enregistrées. enregistrées. Tous les secteurs, toutes nos régions sont touchées. Un record, hélas. L'année 2025 ne semble pas en mesure de corriger cette implacable réalité. 250 000 emplois sont menacées. Et l'annonce de la direction d'ArcelorMittal de 600 licenciements vient encore assombrir le tableau. En Loire-Atlantique, comme sur l'ensemble des territoires concernés, c'est là stupeur. Prendre la décision de licencier 600 salariés après avoir bénéficié de 298 millions de subventions en 2023, puis s'être vu promettre des aides à la hauteur de 850 millions d'euros pour décarboner son activité, c'est incompréhensible pour l'ensemble de nos concitoyens. ArcelorMittal vient s'ajouter à l'inquiétante Litani Michelin-Vancorex-Istovie, générale électrique chez moi encore. La liste n'est hélas pas exhaustive. Certes, les déclarations d'administration de Trump viennent compliquer une situation économique internationale, particulièrement incertaine comme cela a été dit. Mais ces aléas ne peuvent à eux seuls expliquer la fragilisation de notre tissu économique et industriel. L'absence de vision, le manque de planification y sont pour beaucoup. L'objectif de souveraineté industrielle ne peut pas se réduire à la distribution de subventions sans stratégie de sauvegarde et de structuration. Il est plus que temps que l'État s'empare de ce sujet à bras le corps pour initier une réelle politique de développement économique et industriel en en partenariat avec nos territoires et nos représentants européens. Ayons une pensée particulière pour tous les salariés de notre pays qui voient leur avenir et celui de leurs familles. plonger dans l'incertitude sans oublier les territoires qui ne sortent jamais indemne Je me demande donc à quand une planification pour garantir à nos concitoyens, à notre République la souveraineté économique et industrielle que nous sommes en droit d'attendre, et s'agissant d'ArcelorMittal, qu'envisagez-vous de faire Madame la Ministre ? Merci cher collègue, la parole est à Madame la Ministre pour deux minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Philippe Concevalet. Nous avons effectivement pris connaissance des annonces faites par ArcelorMittal concernant le site de Dunkerque dans un contexte de crise sans précédent qui touche à la sidérurgie européenne notamment dû à des surcapacités mondiales et nous ne pouvons que regretter cette décision. Pour autant, en ce qui concerne cette filière sidérurgique, les difficultés datent de plusieurs années. Vous le savez, entre 2018 et 2023, la production européenne a baissé de 20% et en 2024, la demande sur le marché européen a été affaiblit, ce qui crée un certain nombre de surcapacités actuellement. Le plan d'ArcelorMittal concerne tous les sites européens et ne vise pas uniquement et spécifiquement les sites français. Arcelor soutient que ces annonces sont assorties à un objectif prioritaire de restauration de la compétitivité du groupe. Aucun des sites français n'est menacé de fermeture à court terme. C'est important de le rappeler. Il n'y a pas de fermeture à court terme qui est envisagée. Nous serons particulièrement vigilants sur ce point. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracchi, a eu l'occasion de le redire. La France est très mobilisée au niveau européen pour obtenir des mesures fortes de protection du marché de l'acier afin de restaurer une concurrence royale en Europe. Avec huit autres Etats membres, la France a d'ailleurs fait des propositions ambitieuses à la Commission qui se sont traduites par un plan d'action présenté le 19 mars dernier et un premier renforcement des mesures de défense commerciale au 1er avril 2025. Un nouvel instrument de protection commerciale doit être proposé. au plus vite par la Commission, et la France plaide pour qu'il soit le plus ambitieux possible afin de maintenir l'industrie sidérurgique européenne. L'État sera vigilant, très vigilant, quant à la mise en œuvre des annonces par ArcelorMittal, notamment en matière de reclassement des salariés, concernés pour lesquels j'ai également une pensée, et poursuit les discussions avec le groupe pour la confirmation rapide de projets de décarbonation de de Dunkerque et Faust, décarbonation auxquels l'entreprise ArcelorMittal s'est engagée. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Pierre-Antoine Lévy du groupe Union Centriste. Pour deux minutes, c'est à vous chers collègues. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président de la délégation aux entreprises, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaite attirer votre attention sur l'impact dévastateur des retards de paiement dans l'inquiétant de progression des défaillances entreprises. Le rapport remis le 23 avril dernier par les médiateurs Frédéric Wynowski et Pierre Pélousset dresse un constat alarmant. Les retards de paiement à Interentreprise ont atteint un prêt de 14 jours fin 2024, privant non TPE et PME de 15 milliards d'euros de trésorerie. Cette situation est d'autant plus préoccupante que nous traversons une période de croissance ralentie avec seulement 0,9% prévu en 2025, selon la Banque de France. Les chiffres sont parlants. 20% des TPE et 9% des PME présentent des capitaux propres négatifs, témoignant d'une fragilité structurelle inquiétante de notre tissu économique. Dans ce contexte, les retards de paiement constituent souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase menant à la défaillance. Le rapport cite également le frein culturel issu de la honte de l'échec qui conduit à une situation de déni aggravée par l'absence d'informations prévisionnelles de trésorerie. les outils d'aide aux entreprises sont souvent mis en œuvre par des structures qui effraient les chefs d'entreprise comme les tribunaux de commerce, perçus à tort uniquement comme des instances de sanctions et de liquidation. Madame la Ministre, face à cette situation, je souhaiterais connaître votre position sur trois recommandations majeures du rapport. Premièrement, envisagez-vous de modifier le régime des sanctions pour retard de paiement en calculant les amendes en pourcentage de chiffre d'affaires plutôt qu'avec un plafond de 2 millions d'euros manifestement insuffisant pour dissuader les grandes entreprises. Deuxièmement, comment comptez-vous mettre en œuvre la création d'équipes territoriales animées au niveau régional pour fédérer les acteurs publics et privés autour de la prévention des difficultés ? Enfin, la recommandation concernant les formations systématiques des entreprises sur les dispositifs d'aide disponibles, notamment par les experts comptables, me semble cruciale. Comment entendez-vous soutenir cette démarche, notamment pour les TPE-PME, qui n'ont pas les ressources suffisantes pour payer des prestations de conseils ? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Pierre-Antoine Lévy. Vous évoquez un sujet important qui effectivement est une préoccupation quotidienne des entreprises, en particulier les PME et les TPE qui sont les dernières entreprises en bout de chaîne. Les retards de paiement aujourd'hui sont évalués à 15 milliards d'euros de trésorerie dont nos PME et nos TPE manquent et c'est une vraie question de justice économique entre les entreprises privées, quelle que soit leur taille. Structurellement, deux facteurs devraient réduire les délais de paiement à terme. la mise en place progressive de la facturation électronique qui contribuera à une meilleure maîtrise des délais de paiement et l'inclusion depuis 2022 des comportements de paiement dans la quotation des entreprises par la Banque de France. Au demeurant, vous avez raison, la situation législative actuellement n'est pas satisfaisante puisque même si des sanctions existent, qui sont plafonnées à 2 millions d'euros et 4 millions en cas de récidive, le dispositif ne fonctionne pas bien puisque nous avons un certain nombre d'infractions. Je veux d'ailleurs saluer les travaux de la DGCCRF en la matière puisqu'en 2024, 11 amendes supérieures à 1 million d'euros ont été prononcées et nous avons d'ailleurs abordé cette question avec la directrice Sarah Lacoch ce matin et Eric Lombard puisque nous étions dans un site de la DGCCRF sur ce sujet. Nous avons abordé cette question avec le président de la délégation et à un travail en commun pour préparer un texte législatif et t'engager. Le deuxième point que vous évoquez c'est comment organiser une meilleure prévention. Je pense qu'effectivement il nous faut améliorer la lisibilité et faire en sorte d'avoir un point, un guichet unique, une porte d'entrée unique pour les entreprises qui sont en difficulté, je dirais pour les difficultés des entreprises avant même que les entreprises sont en difficulté. Troisième point que vous évoquez, comment mieux accompagner les entreprises. Je pense qu'il faut que nous ayons une charte d'un certain nombre d'acteurs à travers les chambres consulaires, les organisations professionnelles des fédérations, des acteurs privés comme les experts comptables que vous avez évoqué pour améliorer La parole pour améliorer La parole est est à Denis Bouad du groupe socialiste, écologiste et républicain pour deux minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la délégation aux entreprises, mes chers collègues. Je ne pouvais pas participer à ce débat sans vous parler du coup dur qui frappe mon département ces derniers jours. L'annonce de la fermeture de la verrerie de Vergès constitue un véritable honte de choc pour notre territoire. 164 familles sont aujourd'hui dans la détresse. Nous devons garder à l'esprit l'impact de ces de ces événements sur les fermilles qui voient du jour au lendemain leur projet d'avenir remis en cause. Sans repreneur dans les prochains mois, la verrerie de Vergette devra fermer. Alors que 70% de ses commandes sont de son principal client et également voisin direct, il suffit de traverser la route, l'usine Perrier. Cela reprenanterait un non-sens écologique, une perte irréversible pour l'économie et l'ensemble du territoire. La commune de Vergès et l'ensemble des collectivités sont pleinement mobilisées aux côtés des salariés. Mais aujourd'hui, un engagement fort de l'État semble indispensable pour permettre le maintien de cet outil de production. Madame la Ministre, c'est toute une histoire qui a besoin de se sentir soutenue. Nous ne pourrons pas laisser sacrifier la verrerie de Vergès à ses salariés sur l'autel du profit et des stratégies financières. Avec 7% de résultats, comment accepter la fermeture de ce site ? La protection de notre souveraineté industrielle commence par la préservation des emplois industriels existants. On ne peut pas parler de manière crédible de re-industrialisation française face à des salariés qui voient fermer leur usine où ils ont travaillé toute leur vie, parfois de père en fils. Madame la Ministre, comment votre gouvernement compte-t-il s'engager afin de défendre le maintien de ces sites de production, de ces emplois industriels aujourd'hui menacés à Vergès comme ailleurs sur le territoire national ? Merci, cher collègue. La parole est à Madame la Ministre pour deux minutes. Merci, Monsieur le Président. Le sénateur, cette question de l'usine de Verri et de Vergès a déjà été évoquée à travers une question précédente. de noter effectivement un déclin structurel au travers deux marchés clés que sont celui du vin avec une baisse structurelle de consommation qui a entraîné une diminution effectivement. de l'utilisation d'un certain nombre de verres et également sur la bière avec une baisse de consommation et concurrence avec avec l'aluminium. Nous regrettons bien évidemment cette décision de l'entreprise de procéder à ce projet de réorganisation qui s'inscrit dans un contexte économique et financier difficile lié à cette baisse structurelle de la consommation. Sur l'ensemble de ces points, Le gouvernement et les services de l'État sont déjà particulièrement mobilisés et le resteront le temps nécessaire. Un suivi territorial est actuellement initié par le Préfet du Gard et il y associe d'ailleurs l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et politiques du territoire, comme cela se fait dans un certain nombre nombre de situations de même nature. Un suivi identique est instauré dans un grand nombre de situations. À ce jour, plusieurs acteurs ont été mobilisés au travers le service de l'État, la préfecture, la sous-préfecture, le CRP, la DETS du Gard et un certain nombre d'acteurs économiques locaux que sont les agences de développement économique local, notamment celles du conseil régional, des chambres consulaires. Il nous faut effectivement tout mettre en œuvre pour trouver un repreneur et que les salariés puissent retrouver un emploi. En tout cas, le gouvernement est engagé en ce sens. Madame la Ministre, j'entends votre réponse, mais elle ne correspond pas du tout à la question. Je regrette, mais le principal client de la verrerie du Languedoc, c'est la Source Perrier, qui a le même vendu la verrerie, il y a quelques dizaines d'années, pour l'Euro Symbolique. Et aujourd'hui, cette fermeture intervient sur un territoire où la production c'est 70% pour périller, 30% pour les bières. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout sur le problème de viticulture. Alors effectivement, peut-être qu'avec les aides qu'on a apportées, il faudrait-il regarder de près. Merci, Merci, cher collègue. Madame la Ministre, est-ce que vous souhaitez utiliser la réplique ? Non. La parole est à madame Anne-Marie Nedelec du groupe Les Républicains, pour deux minutes. C'est à vous, cher collègue. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'AGS, le régime de garantie des salaires, joue un rôle essentiel d'amortisseur social en avançant le versement des créances salariales dues aux employés lorsque leur entreprise est en procédure collective. Ce mécanisme, financé par les employeurs, représente un filet de sécurité indispensable afin que les défaillances d'entreprises ne se traduisent pas par une précarisation brutale des salariés concernés. La situation économique dans laquelle nous nous trouvons actuellement pèse fortement sur le régime, avec des montants record d'avances versés ces deux dernières années, ce qui a conduit la gouvernance à augmenter par deux fois le taux de cotisation en 2024. À ces difficultés conjoncturelles s'ajoute l'impact de jurisprudence récente de la Cour de cassation qui ont eu pour effet d'étendre progressivement le périmètre de la garantie sur des sommes de nature indemnitaire, s'éloignant ainsi de la mission première de l'AGS qui est de couvrir les créances relatives à la protection de la rémunération. Cela remet en cause la capacité du régime à recouvrer efficacement les fonds avancés aux salariés, or cette capacité à recouvrer, qui est liée pour l'essentiel au statut de créancier prioritaire, est indispensable afin d'assurer l'équilibre financier du régime. Dans ce contexte instable, pouvez-vous nous préciser, Madame la Ministre, les garanties que peut apporter le gouvernement quant à la sécurisation du régime de garantie des salaires ? Pouvez-vous nous confirmer que ce sujet, primordial pour les salariés et les entreprises de notre pays, a bien été identifié par vos services et ceux des autres ministères compétents ? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice Anne-Marie Nedelek, vous avez raison. Le dispositif AGS est un dispositif qui est très utile et qui participe à garantir le paiement des sommes dues aux salariés lorsque notamment deux conditions sont réunies. sont réunies. Lorsque l'employeur est en procédure de sauvegarde de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire et lorsque l'employeur n'a pas les fonds disponibles pour régler les salariés et en tout cas c'est l'objectif initial et premier des AGS. Ce régime permet aux salariés le paiement dans des délais qui sont encadrés de sommes qui leur sont dues. Et d'un point de vue financier, la GS n'a jamais fait faillir et a toujours réussi à assurer sa mission malgré les crises. Et il y a eu quelquefois un certain nombre de situations très différentes avec effectivement des creux et des vagues. Ce fut à à nouveau le cas en 2024 avec 2,13 milliards d'euros d'avance, le plus haut niveau de dépenses depuis 2014. Pour faire face à la dégradation de la conjoncture à la hausse des défaillances, la GS a effectivement relevé ses taux et vous l'avez souligné. Par ailleurs, la GS a conclu le 25 juin 2024 un accord avec les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires dont les effets sur les ressources du régime sont notables. Au premier trimestre 2025, 157,6 millions d'euros ont ainsi été récupéré plus de 53,2% par rapport au premier trimestre 2024 et de même 607 millions ont été récupérés en 2024 par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, plus 72% par rapport à 2023. Donc il y a deux types de rentrées au niveau des AGS, les taux et effectivement ce que récupèrent également les mandataires judiciaires ou les administrateurs judiciaires. Enfin, l'AGS peut recourir à des lignes de prêts auprès des banques en dernier recours, ce qui n'est jamais arrivé. C'est une piste, mais en tout cas, ce n'est pas forcément celle que nous privilégions. Le gouvernement est très attaché à ce régime. Nous sommes vigilants et nous continuerons de suivre ces évolutions de prêts dans les prochains mois, notamment en lien avec avec le ministère du Travail pour répondre de manière précise à votre question. mission première, parce qu'on ne peut pas tout demander tout le temps à l'entreprise. Elles ne sont pas toutes cotées aux 440 d'ailleurs. Et avant de distribuer la richesse, il faut d'abord se donner, et surtout de nos entreprises, les moyens de la créer. Merci, chers Madame la Ministre, est-ce que vous voulez utiliser la réplique ? merci Monsieur le Président. Vous dire que je partage votre vision, vos remarques et en tout cas le gouvernement est très attentif à effectivement ce que l'objectif initial premier de l'AGS qui est de garantir le salaire en cas de défaillance de l'entreprise soit l'élément premier premier et qui doit bien entendu être respecté. Merci Monsieur le Président, merci au Président de la délégation aux entreprises pour l'organisation de ce débat. De nombreux collègues l'ont dit, Madame la Ministre, les défaillances sont en hausse notable. Nous pouvons vérifier dans les tribunaux de commerce de mon département à Vannes et à Lorient qu'il s'agisse des redressements judiciaires ou des liquidations judiciaires quand nous comparons 2024 à 2023. Au-delà, c'est l'emploi menacé parce que ce sont principalement les PMEETI qui sont visés entre 9 et 4 999 salariés, plus 60% en 2024 par rapport à la période de 2017-2019 quand les TPE ne connaissent une hausse que de 16%. Trésorier en baisse, carnet de commande en baisse, stock en hausse dans l'industrie. crise structurelle dans le bâtiment, un climat anxiogène et de latentisme qui se généralisent à la faveur du cycle électoral et des conséquences très directes, Madame la Ministre, des coupes budgétaires que vous avez imposées avec votre gouvernement aux collectivités. J'en viens à l'objet de ma question. S'agissant de la commande publique, le Sénat a lancé une commission d'enquête à l'initiative du groupe Les Indépendants. Nous disons au bas mot ces 170 milliards d'euros par an qui sont mobilisés par les pouvoirs publics, mais en réalité c'est sans doute beaucoup plus. Un rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne estime à peu près 14% la part de la commande publique dans le PIB de notre continent, ce qui nous amènerait à 300 voire 400 milliards d'euros. l'effet est massif. dans le soutien à nos entreprises, nos TPE, nos PME. Et quand on regarde le soutien aux entreprises en difficulté, on a parlé des fonderies de Bretagne, et bien là aussi les collectivités sont au rendez-vous, que ce soit l'Orient en agglomération, la région Bretagne, pour l'aide aussi à la croissance des entreprises qui veulent évoluer en ETI. Et donc pour tout cela, Madame la Ministre, les collectivités ont besoin de soutien, de visibilité, de moyens. Quelles réponses leur apportez-vous ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre, vous avez deux minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Simon Luzonat. Vous avez évoqué plusieurs points. Le premier, vous avez commencé par la commande publique et l'importance de la commande publique en rappelant le montant 170 milliards d'euros. C'est un montant important. Vous évoquiez même celui qui était évoqué au travers le pourcentage du PIB par la cour des comptes. et c'est un soutien important au monde économique et dans ce cadre pour soutenir et plus particulièrement nos TPE, nos PME. Il est important de simplifier l'accès à la commande publique, en tout cas je me réjouis qu'un certain nombre de mesures soit retenue en ce sens dans le projet de loi simplification de la vie économique. Vous m'interrogez ensuite sur finalement la lisibilité et la visibilité dont ont besoin les collectivités territoriales pour s'engager dans un certain nombre d'infrastructures. Je note qu'aujourd'hui les chantiers, les travaux qui sont lancés par les collectivités sont très importants. J'en veux pour preuve les demandes qui sont effectuées auprès des départements dans le cadre notamment des demandes de DETR, des demandes de DECIL. L'ensemble des préfets nous indique aujourd'hui que les demandes sont très importantes donc c'est révélateur en tout cas d'un engagement très fort qu'ont les collectivités pour s'engager dans les infrastructures. Au demeurant Pour une collectivité, il faut avoir plus d'attention que pour les autres. Je pense que c'est la situation des départements qui aujourd'hui se trouvent véritablement en difficulté, notamment compte tenu d'un effet de levier, de financement d'un certain nombre de mécanismes en matière sociale et d'une diminution de ressources. Je pense notamment à tout ce qui est des MTO. Je pense que nous partageons tous et à un certain nombre de rapports d'ailleurs. partagent cette attention particulière en ce qui concerne les départements. Le gouvernement est pleinement engagé. La ministre Catherine Vautrin a d'ailleurs reçu dans ce sens un certain nombre d'acteurs des départements il y a quelques jours. Merci Monsieur le Président. Sur la Merci Monsieur le Président. Sur la simplification, nous pouvons être d'accord, mais les collectivités ont besoin de moyens financiers pour investir, pour soutenir l'économie locale. Vous parlez de la DETR, de la DECIL. Là, nous envoyons les conséquences, y compris dans mon département. Oui, les collectivités font des demandes, elles seront loin d'être toutes satisfaites et beaucoup disent qu'en l'absence de soutien, elles retireront leurs projets. Merci Merci cher collègue. Madame la Ministre. merci Monsieur le Président. Juste rappeler que les montants globalement de DVTR et de Décil n'ont pas changé. Les montants de 2025 sont équivalents aux montants de 2024. Je voulais le redire ici parce que, à vous entendre, j'aurais pu avoir le sentiment qu'il y avait une diminution. Ça n'est pas le cas. Chers collègues, vous avez une minute de réplique. Madame la Ministre, même si l'inflation a baissé, elle est toujours là. Et donc oui, sans prendre en compte l'inflation, c'est à peu près stable, mais pas dans mon département par exemple. C'est moins 2 millions d'euros, donc avec des conséquences pour les collectivités, notamment dans les territoires ruraux. C'est 7 milliards d'efforts que vous avez demandé pour cette seule année 2025, avec probablement des coupes qui seront encore plus importantes dans les mois qui viennent, au regard des discussions qui semblent s'amorcer, au regard aussi des coupes supplémentaires que vous opérez dès cette année 2025, et donc les collectivités sont les élus dans leurs annonces, ils suppriment des projets, ils arrêtent des projets, ils annulent des projets, tout niveau de collectivité confondu, quelles que soient les sensibilités politiques des élus et donc il va y avoir des effets en chaîne potentiellement récessifs pour l'économie qui vont toucher tous les territoires toutes les entreprises et donc madame la ministre nous espérons que votre gouvernement retrouvera le sens de la sagesse sur ce sujet particulièrement important pour les collectivités et les entreprises je vous remercie merci cher collègue la parole est à notre collègue madame lauriane josande du groupe les républicains merci monsieur le président madame la ministre les défaillances d'entreprises sont malheureuses sont malheureusement devenues trop fréquentes dans notre pays. Cela a été dit évidemment aujourd'hui et nous remercions effectivement le président de la délégation pour avoir organisé ce débat d'une importance cruciale. Mon département frontalier des Pyrénées-Orientales illustre parfaitement ce phénomène. En effet, on y relève une hausse de 13% de cessation d'activité par rapport à l'année dernière, soit près de quatre points au-dessus du taux national. Les entreprises du BTP sont particulièrement touchées par ce contexte économique. Ainsi, en 2024, près de 25% des injonctions de pays ont été ordonnées chez nous dans le secteur de la construction. Parallèlement, on observe une hausse de 9,6% des créations d'entreprises. Ce taux est supérieur de près d'un point au national. Les entreprises du secteur du bâtiment comme d'autres illustrent donc le caractère volontariste et particulièrement résilient du territoire que je représente. Et cela pourrait en soi nous rassurer. Mais au-delà des chiffres dont on peut faire des moyennes à l'infini, n'oublions jamais que les défaillances des entreprises sont autant de drames humains et de pertes de savoir-faire difficiles remplacer. Dans mon département sinistré, je vois trop de chefs d'entreprise comme celles créées par mon propre père en 1973 qui se battent chaque jour pour survivre et celles qui finissent par par baisser les bras. En effet, ils font énormément de sacrifices mais constatent aussi avec amertume que de l'autre côté de la frontière, les normes, les charges et la considération envers ces créateurs de richesse et d'emploi ne se valent pas. Madame la Ministre, j'ai donc deux questions. Quel levier le gouvernement compte-il utiliser pour aider les secteurs les plus fragilisés comme le BTP ? Dans l'esprit du test PME deuxième question, le gouvernement entend-il prendre en compte l'impact de la situation des entreprises chez nos voisins européens, notamment dans les zones frontalières lorsqu'il envisage de nouvelles mesures ? Je vous remercie.

l'artisanat. J'ai conscience, j'ai eu l'occasion de le dire, que plusieurs secteurs de l'artisanat, notamment le secteur du BTP, sont confrontés à une forte augmentation des défaillances d'entreprises. à la fois à des hausses et des prix des matières premières, à des diminutions aussi d'un certain nombre de projets en matière de logement, d'inflation, de difficultés de recrutement quelquefois ou de problématiques d'approvisionnement. Demorand, je me réjouis, dans certaines zones, effectivement, il y ait des créations d'entreprises. Vous évoquez également la situation particulière de zones frontalières. qui se trouvent effectivement confrontés à des difficultés de concurrence avec des situations où des entreprises n'ont pas les mêmes normes, n'ont pas les mêmes poids d'impôts, n'ont pas les mêmes dispositifs en matière de compétitivité et cela crée effectivement des distorsions qui ne sont pas faciles à vivre. Par rapport à ça, et je répondrai finalement à votre première question, il nous faut faire en sorte que la compétitivité de nos entreprises s'améliore. Et pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, il nous faut à terme diminuer encore les prélèvements obligatoires. Je vous dis encore parce qu'il y en a eu d'engagées, notamment je pense à ce qui concerne la CVAE, mais il nous faut poursuivre Dans ce scénario, il nous faut également avoir une réflexion probablement sur le financement de la protection sociale. Aujourd'hui, toute la protection sociale, enfin une grande partie, doit continuer à être financée sur les revenus du travail. Pour ma part, je pense que non. Il y a un certain nombre de dispositifs en matière de protection sociale qui, effectivement, doit à mon sens reposer sur le travail. C'est tout ce qui concerne le chômage, la retraite, la maladie professionnelle et les accidents du travail. Mais nous avons deux autres branches que sont les familles et la maladie, où nous pouvons avoir une autre réflexion. Sur le test PME, il faudra prendre en compte, effectivement, des entreprises qui sont frontalières, qui doivent être partie de ce panel pour estimer et mettre en œuvre ce test PME. Merci Madame la Ministre. Vous avez 13 secondes. Madame la Ministre, je vous remercie pour votre réponse très complète et effectivement je crois que la piste que vous évoquez en matière de protection sociale est une excellente piste qu'il faut absolument que nous creusions ensemble et notamment nous nous y emploierons si

l'idée c'est d'avoir un panel d'entreprises. Nous avons évoqué plusieurs fois cette question avec le président Ritman. Dans ce panel d'entreprises, les entreprises qui sont concernées finalement par le texte, que ce soit un projet de loi, un arrêté ou un décret en fonction de la nature du thème du texte qui est retenu, qu'un certain nombre d'entreprises puissent effectivement être volontaires pour répondre à l'enjeu. Et dans ce panel d'entreprises, il doit y avoir des petites et des plus grandes entreprises et de tous les secteurs d'activité, de tous les territoires, y compris des zones frontalières. Chers collègues, vous avez une minute si vous le souhaitez. Écoutez, simplement pour dire encore une fois, nous sommes volontaristes, nous l'avons dit, dans notre territoire des Pyrénées-Orientales et je suis sûre que les entreprises de mon territoire seront volontaires pour participer à cette réflexion et mieux à ces mesures correctrices pour un avenir meilleur qui profitera à l'ensemble du secteur du BTP. Mais au-delà, je le crois, j'en suis profondément persuadée en tout cas, donc je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Damien Michelet du groupe Les Républicains pour deux minutes. Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. D'abord remercier le Président de la Délégation aux entreprises pour l'organisation de ce débat qui rappelle que les entreprises ont leur place au Sénat. La question des défaillances qui nous réunit ce soir nous mobilise en tant qu'élu isèreois, et Frédéric Puyssa se joint à moi, on ne peut pas ne pas parler de Vancorax, de Photowatt, de Valeo, ces entreprises iséroises disparues. Et on voit ce soir que nous sommes tous d'accord sur l'objectif contre la disparition des entreprises. Madame la Ministre, les représentants de l'État ont tendance à minimiser les alertes lancées sur le sujet en rétorquant que la création d'entreprises est toujours dynamique. Et nous en sommes d'ailleurs ravis et du coup il y aurait une balance positive. Mais pour autant, il est dangereux de se rassurer ainsi car la disparition des entreprises entraîne la disparition de savoir-faire précieux, de compétences uniques. Elles remettent aussi en cause certaines chaînes de valeurs et peuvent augmenter notre dépendance aux fournisseurs étrangers. Dans le contexte de guerre commerciale que nous connaissons, cette perspective nous oblige à nous mobiliser pour conserver nos entreprises. Or, à côté des défaillances, nous observons un phénomène de disparition des entreprises qui, faute de préparation insuffisante en amont, n'ont pas pu être transmises. Dans son dernier rapport sur la transmission d'entreprises, la délégation a montré le caractère essentiel du pacte du travail pourtant ignoré de 82% des chefs d'entreprises consultés. Pourtant, ce dispositif permet des transmissions aux familles ou aux salariés. Madame la Ministre, je sais que vous êtes sensible à la question de la transmission d'entreprises. La transmission, c'est de l'emploi, c'est de la valeur ajoutée pour nos territoires, des savoir-faire conservés et puis de la fierté collective. Mais ma question, Madame la Ministre, Le gouvernement va-t-il enfin lancer une campagne d'information auprès des dirigeants de TPE et de PME afin de mieux les sensibiliser à ce sujet et à leur présenter le pacte du trade, qui est une vraie assurance vie à la transmission. Les entreprises les plus modestes en taille sont aussi concernées que les autres, mais elles manquent évidemment d'accompagnement et de sensibilisation. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Damien Michelet. Vous avez évoqué la défaillance des entreprises. Les créations ont une balance positive mais effectivement il faut être très vigilant par rapport à cette balance positive parce qu'on a des créations d'entreprises, j'ai eu l'occasion de le dire, avec beaucoup de de très petites entreprises. Je rappelle qu'en 2024 c'est 1 million 100 mille entreprises qui se sont créées dont 700 mille micro-entreprises. Et de l'autre côté nous avons effectivement des défaillances et au-delà des défaillances vous évoquez le nombre d'entreprises qui arrêtent, qui cessent sans que pour autant il y ait des défaillances. Si nous avons eu 66 000 défaillances en 2024, c'est 165 000 entreprises qui ont arrêté à côté en sus des défaillances. Donc vous avez raison, il faut effectivement se préoccuper de tout ce qui concerne la transmission et la reprise. Je veux juste souligner que le pacte du trade est un excellent pacte qu'il nous faut bien entendu maintenir parce qu'il participe à une transmission des entreprises dans le secteur familial le plus souvent. et que ceci permet d'économiser un certain nombre de de droits qui permet à l'entreprise de pouvoir se développer, continuer à investir, à innover et finalement réussir sa transmission. Je note d'ailleurs qu'une proposition de loi pour une politique de la transmission a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale le 4 février dernier pour faire évoluer le pacte du trade dans un pacte du trade long terme avec une augmentation du seuil d'exonération mais un engagement qui devrait être pris dans la proposition de loi d'aller au-delà de la période de 8 ans, d'aller jusqu'à 10 ans. Vous dire que sur cette question de transmission et reprise des entreprises, je m'en préoccupe parce que nous savons que c'est 700 000 entreprises qui vont cesser dans les 10 ans qui viennent. On évalue à peu près à ça, il y a des chiffres un petit peu différents. Et aujourd'hui nous avons une entreprise sur deux qui n'est pas reprise. Une entreprise sur deux. Donc c'est relativement important. Je vais lancer, j'ai eu l'occasion d'ouvrir auprès du Président de la délégation sénatoriale, des assises de la transmission reprise pour mettre autour de la table l'ensemble des partis prenants, les chambres consulaires, les organisations professionnelles, les acteurs, les parlementaires, pour que nous puissions faire émerger un certain nombre de propositions. Merci Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Elsie Joseph du groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais aborder le sujet du suivi de l'impact des défaillances d'entreprises. Ce suivi peut être complexe parce qu'il varie selon plusieurs critères, trois critères. Tout d'abord le critère sectoriel puisque, d'après les chiffres de l'AGS, 6 secteurs concentrent plus de 80% des salariés bénéficiaires de la garantie des salaires. L'industrie, la construction et les services aux entreprises sont les plus touchés. Mais il y a aussi des progressions inquiétantes comme celle du secteur agricole qui représente un volume moindre mais a connu en 2024 la plus forte hausse de défaillance avec plus de 37%. Ensuite, il existe le critère géographique. Selon celui-ci, c'est sans surprise l'Île-de-France qui concentre 28% du total des montants versés par la GS. Enfin, il existe évidemment un critère stratégique. Certaines entreprises peuvent être clés pour l'indépendance de la production française ou pour la conservation d'un savoir-faire. Madame la ministre, compte tenu de la multiplicité des critères et des données, comment votre ministère et plus généralement le gouvernement pilotent-ils le suivi des défaillances d'entreprises ? Quels sont les indicateurs clés pour lancer une alerte ? Comment s'organiser les services de l'Etat pour repérer les défaillances les plus inquiétantes pour notre économie ? Elles le sont toutes du point de vue de l'emploi, mais pas forcément d'un point de vue de la souveraineté économique par exemple. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice Else-Joseph. Vous avez raison, il y a un certain nombre d'indicateurs clés qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations sur les défaillances d'entreprises, de manière générale ensuite, par secteur d'activité, par région, par nature d'entreprise, notamment en fonction de l'effectif. L'ensemble de ces éléments nous permet d'avoir des informations d'ailleurs dont en règle générale les parlementaires sont assez friands parce que ça nous permet aussi de préparer, de conduire des politiques publiques pour à la fois essayer d'éviter bien entendu des défaillances parce que je crois qu'avant d'accompagner ou de soutenir ou d'être en appui aux défaillances l'objet c'est quand même d'éviter qu'il y ait un certain nombre de défaillances. Par rapport à ces situations il n'en demeure pas moins que la prévention est très importante et qu'il y a un projet informatique qui est intitulé Signeaux faibles, qui est un projet qui est géré par une start-up d'État sous la tutelle de la direction numérique des entreprises, qui a été conçu pour répondre à l'urgence de la crise du Covid-19 et qui finalement a été pérennisé. Et grâce à cet outil informatique, Avec cet outil informatique, c'est grâce à cet outil informatique que les comités départementaux détectent un certain nombre d'entreprises au travers des alertes et cela permet un accompagnement en préinvention et nous savons que tout ce qui participe à un accompagnement permet quelquefois d'ailleurs d'accompagner les entreprises vers les procédures amiables avant de rentrer dans les procédures et quand c'est accompagné dans des procédures amiable 70% des entreprises ne vont pas vers les procédures collectives. Voilà donc ces éléments permettent de nourrir je dirais les politiques publiques qui sont conduites et d'améliorer effectivement tout ce qui participe à l'accompagnement au soutien.

des AGS, souvent d'ailleurs parce qu'on a des entreprises en difficulté dans le secteur de la fonderie et de la métallurgie, ce qui remonte du terrain, c'est qu'on dénonce pardon, la multiplicité des intervenants, trop de comités, trop d'acteurs, trop de dispersions. Donc c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez redit tout de suite, comment mieux intervenir en amont. Par exemple, moi ce qui m'a remontée, c'est que par exemple le tribunal de commerce peut conseiller mais le mot tribunal, en tout cas c'est le cas dans mon département, fait souvent peur. Donc il est peut-être pour moi impératif d'avoir un guichet unique et en tout cas plus de simplicité et plus d'informations données à toutes les parties prenantes. Merci. Merci cher collègue Madame la Ministre, vous avez une minute. Oui, merci Monsieur le Président. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on a une difficulté de lisibilité qui ne permet pas forcément aux chefs d'entreprise de frapper à la bonne porte. Et c'est un sujet d'ailleurs qui a été évoqué dans le rapport de la Cour des comptes, qui a été remis en juin en juin dernier, qui a été évoqué également dans un rapport que m'ont remis le médiateur du crédit, le médiateur des entreprises. quelques jours. J'ai eu l'occasion d'évoquer ça également la semaine dernière dans la Loire. Je pense qu'il nous faut aller vers la réflexion d'une porte unique. Je pense très sincèrement qu'aujourd'hui l'acteur qui pourrait être la porte unique et le conseiller des et le conseiller départemental aux entreprises en difficulté dit autrement CDED qui peut être la porte d'entrée et qui après peut orienter vers les CRI pour les entreprises de plus de 400 salariés vers le CRP pour les entreprises de 50 à 400 salariés je crois que c'est important d'avoir effectivement une porte d'entrée qui pourrait être ce conseiller départemental en tout cas je vais continuer à travailler sur ce sujet Merci madame la madame la ministre, madame la ministre, chers collègues, vous avez une minute ? Juste une seconde, merci pour ces éléments, je pense que ça va rassurer mon territoire parce qu'en amont évidemment de ce débat, j'ai consulté beaucoup et franchement on n'a que des ressentis, on a l'évolution des carnets de commandes, on ne sait pas qui s'adresser et je pense que c'est une bonne nouvelle et on faudra communiquer sur ce sujet, merci. Merci chers collègues, la parole est à notre collègue madame Sylvie Valente-Lehir du groupe Les Républicains pour deux minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Panhard, Citroën, Peugeot, Renault sont devenus des noms synonymes de notre histoire industrielle et automobile française au cours du XXe siècle. L'automobile a transformé notre quotidien et façonné nos territoires. L'exemple de Peugeot à Sochaux l'illustre parfaitement, tout comme celui de Michelin, A Clermont-Ferrand. Or, ce que nous imaginions impensable est en train de survenir. Notre filière automobile et ses sous-traitants sont purement et simplement menacés de disparition. Les causes sont plurielles. Concurrence étrangère, choix industriel erroné, décision politique inconsidérée. Les chiffres sont impressionnants. 149 000 entreprises, 990 000 emplois directs et indirects, 155 milliards de chiffres d'affaires, 6 milliards d'euros investis chaque année dans la recherche et développement selon les sources officielles du ministère. Prenons pour exemple la ville de Meru. dans le département de l'Oise dont le projet de PSE affectant le centre technique Forvia a entraîné en novembre dernier 102 postes supprimés dans le service recherche et développement. Ce fut un cataclysme pour cette ville de près de 15 000 habitants. Traumatisme d'autant plus fort qu'en juillet 2020, le ministre de l'économie, monsieur Bruno Le Maire, était venu sur place pour parler verdissement et relance de l'économie. D'autre part, les dernières annonces du président des Etats-Unis Donald Trump à travers une augmentation sans précédent des droits de douane viennent noircir davantage encore un tableau déjà sombre. Comment être conscient de cette situation et laisser faire ? et laissons faire. Par conséquent, alors que le libre-échange devient de plus en plus théorique en raison de la montée en puissance de nouveaux acteurs tels que la Chine qui subventionne allègrement ses constructeurs, nous, Européens, nous refusons d'accompagner les nôtres. Pire encore, nous leur imposons un calendrier seul et contre toute réalité de fin de vente des véhicules thermiques en Europe à l'échéance 2035. C'est pourquoi dans ce contexte, sans modification des règles en vigueur, nous nous condamnons à vivre et revivre les mêmes scénarios qu'à Meru.

la situation d'une entreprise de votre territoire qui finalement subit l'impact de toute la filière automobile. Vous rappelez que les ventes de véhicules en France sont structurellement en baisse depuis les années 2000, mais la chute est aussi très récente avec près de moins 25% d'immatriculation par rapport à 2019, avec des impacts aussi différents, puisqu'il a été fait le choix de sortir du véhicule thermique en 2019. 35 et que nous sommes aujourd'hui au milieu du guet puisque les constructeurs automobiles ont investi pour transformer leur industrie. Des bornes de recharge commencent à être déployées, les utilisateurs de véhicules électrique commence à être de plus en plus nombreux et cette technologie va continuer à s'imposer sans aucun doute dans les années qui viennent. Au demeurant chantant, l'industrie l'industrie automobile est fortement percutée et que certaines entreprises ont annoncé La suppression, c'est le cas de Forvia qui a annoncé la suppression de 10 000 emplois en Europe du fait du contexte du marché automobile. Il faudra être attentif à tout ce qui concerne les propositions de reclassement pour faire en sorte que ces 10 000 emplois puissent être accompagnés, que ces emplois supprimés puissent être accompagnés. Il faut également soutenir la filière automobile française ou la filière automobile européenne, mais je pense à la filière automobile française pour que celle-ci puisse se transformer. Nous devons continuer à l'accompagner. Ça a été le cas d'un certain nombre de dispositifs France Relance, France 2030, pour accompagner l'industrie. C'est ce que nous faisons encore au travers un certain nombre de situations. Je rappelle que France 2030, c'est 54 milliards d'euros qu'on est engagé pour soutenir l'industrie à se rénover, à préparer, je dirais, le futur. Merci Madame la Ministre. Pour conclure ce débat, la parole est à Christian Klinger de la délégation aux entreprises pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la délégation aux entreprises, Mes chers collègues, Des débats comme celui d'aujourd'hui sont riches et démontrent l'utilité de la délégation aux entreprises qui a pour mission d'aborder les sujets de façon transversale en complément des travaux des commissions permanentes. Vous l'avez vu, à travers les questions de nos collègues, Madame la Ministre, seule une approche globale permettra d'aborder de façon pertinente la question des défaillances d'entreprises. la simplification des normes, la concurrence européenne et internationale, le développement des PME et des ETI, la transmission des entreprises, les retards de paiement, le développement des compétences ou la viabilité financière de l'AGS. Il n'est pas possible de s'attaquer au sujet des défaillances à travers un prisme unique. J'aurais pu rajouter à cette liste d'ailleurs la question du foncier économique puisque j'ai été l'auteur avec mon collègue Michel Masset d'un rapport de la délégation sur ce sujet pour lequel nous aurions tant de progrès à accomplir. Pour ce sujet d'ailleurs, comme pour tous ceux qui concernent les entreprises, il y a un réel problème de délai. Les décisions politiques, devant apporter des solutions, sont prises dans des délais beaucoup trop longs. Les présidents des organisations patronales nous l'ont dit cet après-midi lors d'une table ronde. Le temps des mesures politiques est trop long, en total décalage avec celui de la vie économique. L'action publique doit impérativement gagner en agilité. Tous les sujets que la délégation analyse depuis sa création et pour lesquels elle propose des solutions très concrètes doivent être traités si l'on veut éviter que les chiffres des défaillances ne repartent fortement à la hausse dans le contexte actuel de guerre commerciale. Et ils doivent s'accompagner d'une véritable stratégie de soutien à la compétitivité des entreprises, comme l'a rappelé le président de la délégation, Olivier Ritman. Tout ce que nous nous sommes dit au cours de ce débat n'aura de sens que si nous prenons conscience de l'impact de nos décisions, notamment lors des arbitrages budgétaires à venir. J'insiste sur la nécessité de porter des réformes structurelles visant à réduire la dépense publique, plutôt que de miser sur une contribution toujours plus importante des entreprises. Dans une récente tribune, le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourc, nous interpelle en débutant ses propos ainsi. Il est honnêtement dur d'être européen en ce moment, regrettant que l'Europe ne soit un prédateur en rien et doivent subir les attaques des États-Unis et de l'Asie. Il ajoute « comme on le fait avec les faibles, on nous piétine des deux côtés ». Comme lui, je souhaiterais redire que nous devons être courageux. Cette vision d'une Europe qui se tire une balle dans le pied, beaucoup de dirigeants la partagent encore davantage pour la France, dont la fiscalité et les impôts de production en particulier constituent un handicap pour les entreprises françaises. Alors, ayons le courage de continuer ce débat, dans les mois qui viennent pour aborder la question du projet de loi de finances pour 2026 avec pragmatisme et clairvoyance. La souffrance des territoires touchés par les défaillances d'entreprise, Madame la Ministre, vous l'avez entendu par le truchement des questions de mes collègues sénateurs. Ce sont autant de drames que nous souhaitons tous éviter. Nous avons compris que vous partagez la même préoccupation, Madame la Ministre. Comme vous le disiez en introduction, c'est la base d'un dialogue. Et les échanges de ce soir constituent donc une première étape dont nous pouvons nous réjouir. Mais la suite à donner requiert une mobilisation urgente sur tous les fronts. Nous continuerons à rappeler les réalités du monde économique et à défendre les mesures qui doivent devenir prioritaires afin que la tendance des défaillances d'entreprises décrites ce soir puisse enfin s'averser. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h40 pour le débat sur les initiatives européennes en matière de simplification et d'allègement de la charge administrative pesant sur les entreprises. La séance est suspendue.